pour objet de créer des postes de magistrats assistant d'autres magistrats. Je considère que, lorsqu'un magistrat sort de l'École nationale de la magistrature, il doit exercer la plénitude de ses fonctions et qu'il ne saurait être magistrat assistant d'un autre magistrat. Mon projet consiste, à l'inverse de ce que propose la commission, à recentrer le magistrat sur le coeur de son office, à l'employer à son juste niveau de compétence et de responsabilité. C'est la raison pour laquelle j'envisage de créer de l'assistance pour les magistrats. Il ne s'agit donc pas du même processus. Le projet de loi de programmation que je vous ai soumis il y a quelques jours crée à cette fin cinquante postes d'assistants de magistrats par an. La deuxième raison pour laquelle je m'oppose au texte de la commission est une raison de fond. La réflexion sur l'ensemble de la problématique liée aux questions qui sont débattues est, me semble-t-il, insuffisamment aboutie. J'ai ainsi été surprise de constater que la

La troisième raison de notre divergence tient à la méthode. La mobilité des magistrats, la durée minimale et maximale de maintien à un poste, la nomination et l'évaluation des chefs de juridiction et de cour sont des questions réellement importantes, que vous avez voulu soulever. Elles rejoignent d'ailleurs les questions relatives au déroulement de carrière et à l'accès aux postes de responsabilité. Toutefois, légiférer immédiatement sur ces sujets-là, sans qu'une large concertation ait été engagée avec les magistrats et leurs représentants syndicaux, serait, selon moi, pour atteindre l'objectif d'amélioration du service public de la justice que nous partageons. Ces points méritent une concertation élargie et spécifique et, le cas échéant, une loi particulière. Je ne suis pas opposée à y travailler. Telles sont les raisons

Les objectifs que cherche à atteindre la commission des lois sont parfaitement louables : il s'agit de limiter un turn-over excessif qui nuirait au bon fonctionnement des juridictions et de garantir l'impartialité objective des juges en ne les laissant pas toute leur vie professionnelle durant sur un même poste. Cependant, je souhaite retirer cette disposition pour les raisons que j'ai évoquées. J'y ajoute une contrainte de gestion. Inscrire dans la loi une durée minimale de trois ans mérite une réflexion approfondie, car la gestion des ressources

amendement vise à supprimer l'institution des durées minimale et maximale d'affectation des magistrats au sein d'une même juridiction. Ce dispositif a été introduit par la commission des lois et reprend les dispositions de l'article 2 de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice que le Sénat a adoptée le 24 octobre 2017. Ces dispositions, d'ailleurs déclinées dans d'autres articles

notamment celui de la mission d'information du Sénat sur le redressement de la justice, rapport qui date du mois d'avril 2017 et qui a fait l'objet de larges concertations, à la fois auprès des magistrats, de leurs syndicats représentatifs et, naturellement, de toutes les personnes susceptibles de donner un point de vue sur ce sujet.

Néanmoins, nous avons l'impression que l'on nous renvoie une nouvelle fois au sixième chantier de la réforme de la justice sur les ressources humaines, dont on nous indique qu'il sera mené dans le cadre de la loi organique qui suivra l'adoption de la loi constitutionnelle réformant le Conseil supérieur de la magistrature. Nous ne savons pas quand

Pourtant, le sujet nous semble urgent. Il peut en outre être traité indépendamment de la réforme du CSM, s'agissant de la modification du statut de la magistrature. Le dernier rapport d'activité du CSM pour l'année 2017 confirme, à cet égard, « le phénomène de mobilité qui caractérise désormais les carrières des magistrats » et fait état de l'examen de 2 856 propositions de nomination du garde des sceaux, soit près de 35 % du corps des magistrats. La mise en place d'une durée minimale d'exercice des fonctions, telle que nous la proposons,

de cette forte mobilité ». Selon ce rapport, celle-ci « rend plus difficile l'investissement des magistrats dans les fonctions et le travail en équipe. Elle peut ralentir la mise en oeuvre des projets de service et de juridiction. Elle peut enfermer certains chefs de juridiction dans une gestion à court terme de la structure qui leur est confiée, faute de prévisibilité sur la composition des équipes. Des mouvements fréquents touchant certaines fonctions de cabinet génèrent des vacances de poste répétées qui nuisent à la célérité du traitement des dossiers. Une forte mobilité plus ou moins subie entraîne des conséquences lourdes sur la vie personnelle et familiale. Elle a une incidence sur le déroulement de la carrière des femmes ». S'agissant de la durée maximale d'exercice des fonctions que nous proposons, le rapport du CSM relève également qu'« il n'existe aucun outil permettant d'identifier les situations de grand immobilisme touchant certaines juridictions, notamment parmi les plus attractives et susceptibles de créer des difficultés au plan déontologique ». Compte tenu de ce contexte largement documenté, nous considérons que l'institution de nouvelles règles constitue un impératif au regard des difficultés de gestion des ressources humaines et, surtout, de leurs conséquences en termes de désorganisation de nos juridictions. Cependant, pour tenir compte des exigences de souplesse de gestion, l'article 1 A prévoit également la possibilité de déroger à ces règles sur avis motivé du CSM. Par ailleurs, nous estimons que ces règles sont conformes aux principes de portée générale définis par la jurisprudence constitutionnelle, et ne portent atteinte ni au principe de l'inamovibilité des magistrats du siège ni à aucun autre principe ou exigence de valeur constitutionnelle. Elles s'appliqueraient à tous les titulaires des fonctions en cause. Les magistrats devront être pleinement informés de la limitation dans le temps de la fonction. Ainsi, en acceptant ces règles, ils auront consenti aux modalités d'affectation prévues par la loi organique. De ce fait, les nouvelles obligations de mobilité et les conséquences qui s'y attachent ne peuvent s'appliquer que dans un délai suffisant pour permettre aux magistrats de prendre connaissance de ces nouvelles règles, qui peuvent impliquer un régime transitoire. C'est la raison pour laquelle l'article 1 A prévoit que les dispositions ne sont applicables qu'aux magistrats nommés à compter du 1 septembre 2019, sauf pour ceux auxquels s'applique le régime transitoire, naturellement.

par la suite des améliorations éventuelles. Enfin, des garanties de nature à concilier les conséquences qui résultent d'une obligation de mobilité avec le principe de l'inamovibilité des magistrats du siège sont également prévues dans le dispositif de l'article 1 B du projet de loi organique.

En conséquence, je souhaite intégrer à l'ordonnance statutaire les fonctions de juge et de vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection. Quel est l'avis de la commission

le magistrat, si son service n'est pas complet, d'apporter un complément de service dans d'autres fonctions, selon ce que lui demandera le président du tribunal.

excessivement l'organisation d'une juridiction, puisque le président du tribunal confiera à ce juge les contentieux qui existent et qui ressortent de son champ de compétences, mais si le service de celui-ci n'est pas complet, il pourra aussi l'affecter à d'autres chambres ou à d'autres sections.

garde des sceaux. La commission a prévu un dispositif permettant au président d'une juridiction de désigner un magistrat du siège ayant prêté serment depuis moins de trois ans pour accorder son concours à un autre magistrat pour la préparation de la décision, lorsque la nature de l'affaire le justifie. Le présent amendement a pour objet de supprimer une telle disposition.

je ne suis pas sûre qu'il soit pertinent d'instituer un tutorat de cette manière. Les équipes autour du magistrat me semblent réellement performantes et sont d'ailleurs souhaitées par tous les magistrats. Il s'agit d'une solution qui est mieux adaptée à la réalité du travail des magistrats que celle que vous proposez.

je suis défavorable à l'instauration

garde des sceaux. L'article 1 introduit par la commission instaure la possibilité de nommer les auditeurs de justice à un premier poste de magistrat du siège

dans le texte par la commission. Sur le fond, l'article 1 prévoit que des auditeurs de justice pourraient être nommés en premier poste auprès d'un magistrat du siège exerçant ses fonctions au sein d'une juridiction qui détient des compétences particulières ou au sein d'une juridiction spécialisée. L'objectif est de créer pour les magistrats du siège une sorte de pôle d'excellence, sur le modèle de ce qui existe déjà pour les magistrats du parquet avec les juridictions interrégionales spécialisées, que l'on appelle plus communément les JIRS. La commission est défavorable

La commission des lois a fixé une durée minimale d'exercice des fonctions de conseiller et d'avocat général référendaire à la Cour de cassation. Ainsi que je l'ai déjà exposé, je suis défavorable à l'instauration dans le à l'instauration dans le statut de la magistrature de délais minimaux d'exercice des fonctions. Cela aboutirait en effet à la suppression d'une indispensable souplesse dans la gestion des ressources humaines. Dans la pratique, d'ailleurs, une durée minimale de trois années est déjà fixée pour les postes de conseiller et d'avocat général référendaires, sauf situations exceptionnelles. Dans

garde des sceaux. La commission a introduit des critères d'appréciation que le Conseil supérieur de la magistrature devrait prendre en considération pour proposer ou donner son avis sur la nomination des chefs de juridiction. dispositif peut paraître légitime, à savoir fixer des critères précis de sélection pour ces postes à haute responsabilité. Cependant, la fixation de tels critères dans une loi organique rigidifierait la procédure de nomination.

est à Mme la garde des sceaux. Monsieur le rapporteur,

garde des sceaux. La commission a fait référence à des critères d'appréciation que le Conseil supérieur de la magistrature devrait prendre en considération

sceaux. Le présent amendement vise à modifier les compétences des magistrats exerçant à titre temporaire. Compte tenu de la création de la fonction de juge des contentieux de la protection et de leur exercice dans les tribunaux de proximité, ces magistrats

Cet amendement a pour objet de créer la fonction de procureur de la République antiterroriste près le tribunal de grande instance de Paris.

la garde des sceaux. Cette disposition transitoire permet aux actuels juges d'instance de continuer à exercer leurs fonctions au sein d'un tribunal de grande instance ou d'une chambre de proximité en qualité de juges des contentieux de la protection.

Cet amendement a pour objet de différer l'entrée en vigueur des articles relatifs à la création des fonctions de juge des contentieux de la protection au 1 janvier 2020.

Le vote, par scrutin public ordinaire, en application de l'article 59 du règlement, aura lieu le même jour, à seize heures, à la suite de la proclamation du scrutin public solennel sur le projet de loi ordinaire. Je n'ai été saisi d'aucune observation sur les conclusions de la conférence des présidents. Elles sont donc adoptées. Voici quel sera l'ordre du jour de